président de cette collectivité. Au contraire, nous souhaitons maintenir le pouvoir de police de la circulation du préfet de département sur ces axes, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur vocation structurante et des enjeux de sécurité. Quel est l'avis de la commission

engagés sur les portions de route inachevées. Cela semble plein de bon sens, mais je veux rassurer notre collègue : les dépenses engagées par l'État seront payées, comme c'est la règle. Par ailleurs, l'article 6 prévoit expressément l'achèvement de toute opération inscrite au

seulement sur la voirie nationale non concédée et sur les voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic du fait de l'instauration d'une écotaxe sur la voirie nationale. Paradoxalement, l'écotaxe proposée ne trouverait donc pas à s'appliquer en Alsace, où l'intégralité de la voirie nationale devrait être transférée au département.

L'accord entre le Gouvernement et les trois collectivités, ainsi que le présent projet de loi, transfèrent à la Collectivité européenne d'Alsace le réseau routier national en Alsace, dont des autoroutes non concédées. À terme, l'eurométropole de Strasbourg pourra également bénéficier, à sa demande, du transfert des portions de voies précitées situées sur son territoire. Ce transfert doit permettre la mise en place d'une régulation du trafic de transit à l'échelle transfrontalière,

les responsables alsaciens demandent la mise en place d'un système similaire sur leur territoire et les plus anciens d'entre nous se souviennent qu'à l'époque un député

cet amendement vise également à compenser la création de cette taxe par un dégrèvement sur la cotisation foncière en faveur de ces dernières. Le sous-amendement

à la future directive Eurovignette, en cours de négociation. La commission a néanmoins considéré que l'habilitation demandée par le Gouvernement à l'article 10 était très floue

du Gouvernement, qui a cru pouvoir régler à l'échelon d'un département toute la problématique liée au trafic nord-sud.

pas difficile d'imaginer que, dans ces conditions, le trafic se déporterait et que les Lorrains, solidairement avec les Alsaciens, devraient pouvoir se protéger ! Je ne comprends pas que l'on ait pu appréhender

malheureuse. Tirant les conclusions de ces expériences, cet amendement prévoit que la taxe sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes sera instaurée à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans.

La commission a souhaité inscrire dans le projet de loi le principe selon lequel les agents non titulaires des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat lors de la fusion des départements et de la reprise des

dans cette base de calcul toutes les dépenses d'investissement qui relèvent de l'exercice ordinaire des responsabilités de l'État en tant que propriétaire des routes, les aménagements de sécurité, de sécurité, mais aussi ceux qui visent à améliorer la fluidité du trafic ou à prévenir des dommages à l'environnement, la réhabilitation d'ouvrages menaçant ruine. La commission a en revanche exclu de la base de calcul les compensations pérennes des dépenses liées à des investissements exceptionnels, c'est-à-dire la construction de voiries nouvelles ou l'élargissement des voiries existantes. La parole est à M.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution imposent au législateur, lorsqu'il transfère aux collectivités des compétences auparavant exercées par l'État, de leur attribuer des ressources correspondant aux charges constatées à la date du transfert.

à M. André Reichardt. Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe d'éligibilité au financement par les contrats de plan État-région des futures opérations routières menées par la Collectivité européenne d'Alsace sur le réseau sur le réseau routier national transféré à compter du 1 janvier 2021, eu égard à leur caractère structurant et à leur rôle de desserte à l'échelle routière européenne.

collègues craignent que, à la suite du transfert de la voirie nationale non concédée au département d'Alsace, celui-ci ait à assumer seul le coût de l'ensemble des travaux sur la voirie transférée. En l'état du droit, rien n'empêche l'État de subventionner des opérations dont le maître d'ouvrage est un département, que ce soit dans le cadre du CPER

après la création de la Collectivité européenne d'Alsace. Cette mesure transitoire prévoit que les actes et délibérations demeurent en vigueur, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace. Ce remplacement devrait intervenir au plus tard le 1janvier 2027. En d'autres termes, pendant une période de six ans, certaines normes adoptées par les anciens départements demeureraient en vigueur jusqu'à leur remplacement. Nous sommes dubitatifs. Cette dérogation vise-t-elle à garantir la continuité du service public et de l'exercice des compétences départementales ?

est à M. le ministre. Par cet amendement, le Gouvernement souhaite rétablir la rédaction initiale de l'alinéa 3 de l'article 8, relatif à l'élection des conseillers départementaux de la Collectivité européenne d'Alsace et par là même supprimer des dispositions relatives à l'élection des conseillers régionaux introduites par la commission des lois. des lois. La commission des lois a supprimé l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour adapter les règles relatives à la composition du collège électoral concourant à l'élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui était prévue à l'article 9

des électeurs du Haut-Rhin habitant dans un canton rattaché au Bas-Rhin seraient appelés à élire un député du Bas-Rhin.

Les alinéas 15 et 16 prévoient de fixer leur nombre à soixante. Il convient en effet que ce nombre soit calculé en fonction des populations actuelles des différentes sections de la région Grand Est, afin de respecter les équilibres démographiques actuels. Le Gouvernement estime cependant que les changements à apporter au code électoral pourront l'être par voie

nombre de cantons des départements est déjà fixé par le code général des collectivités territoriales. Il convenait simplement de l'adapter à la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace. Néanmoins, dès lors que les règles concernant l'élection sénatoriale sont maintenues et fixées dans la loi, la commission émet un avis de sagesse.

je ne sais toujours pas quelle est véritablement la position du Gouvernement à l'égard de l'avis du Conseil d'État

été exprimé. Je remercie tout particulièrement notre rapporteur, Agnès Canayer, pour son excellent travail, pour le compromis qu'elle a su trouver.

Je crois que l'exercice auquel nous nous sommes livrés est assez salutaire, dans la mesure où il nous montre la complexité des débats que nous aurons sur la différenciation.

rédaction qui va aussi loin que possible dans le cadre constitutionnel actuel. Cela dit, j'ai observé que le Gouvernement

les Alsaciens considèrent que ce projet de loi, même amélioré par le Sénat, ne va pas encore suffisamment loin

sur le malheur des autres, ni son développement au détriment de celui des autres ! Cette belle solidarité a permis de trouver un accord quasi je m'en félicite. Nous avons appris les uns des autres. Et animés de cet esprit d'écoute et de compréhension mutuelle, nous construisons de beaux textes. Je regrette cependant

les différentes facettes de cette nouvelle Collectivité européenne d'Alsace. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de mes collègues de la qualité des débats : ceux-ci ont parfois été vifs, voire enflammés,

sans pour autant porter atteinte aux compétences des autres départements de la région Grand Est. Nous avons été attentifs à garantir la volonté et l'accord systématique des départements et de la région, pour